vingts ans, le 27 janvier 1945, les troupes soviétiques libéraient le camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz Birkenau, en Pologne, où plus d’un million de personnes sont mortes. En ce jour de souvenir, le Sénat est associé aux commémorations organisées autour du 80 anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz. Notre collègue Francis Szpiner a représenté ce midi M le président du Sénat à la cérémonie d’hommage en mémoire des victimes de la Shoah qui s’est tenue au mémorial de la Shoah. En fin de journée, notre collègue Jocelyne Guidez assistera au ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe en présence du Premier ministre et de représentants de l’Union des déportés d’Auschwitz. Plus que jamais, nous devons rester vigilants et intraitables face à la résurgence de toutes les formes d’antisémitisme et d’appels à la haine. N’oublions pas. En application de l’article L.O. 153 du code électoral, M. Philippe Tabarot, qui a été nommé membre du Gouvernement, a cessé d’exercer son mandat de sénateur le jeudi 23 janvier 2025 à minuit. Par lettre en date du 27 décembre 2024, le ministère de l’intérieur a fait connaître au président du Sénat qu’en application de l’article L.O. 320 du code électoral, M. Jean Marc Delia a remplacé M. Philippe Tabarot en qualité de sénateur des Alpes Maritimes.

En application de l’article L.O. 320 du code électoral, le mandat sénatorial de Mmes Agnès Canayer et Laurence Garnier a repris le vendredi 24 janvier 2025 à zéro heure. En conséquence, le mandat sénatorial de Mme Virginie Lucot Avril et de M. Maurice Perrion a cessé le jeudi 23 janvier 2025 à minuit. Je salue le retour de nos collègues. J’informe le Sénat qu’ont été publiées des candidatures pour siéger au sein de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ; de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport de la commission d’enquête aux fins d’évaluer les outils de la lutte contre la délinquance financière, la criminalité organisée et le contournement des sanctions internationales, en France et en Europe, et de proposer des mesures face aux nouveaux défis ; de la délégation sénatoriale aux entreprises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

Six ans plus tard, […] nous sommes proches de l’humiliation économique. Le décrochage de l’Europe dans le monde, et de la France en Europe, n’a pas commencé avec cette histoire de, mais l’accélération est vertigineuse après la crise de 2008, le PIB de l’Union européenne était équivalent à celui des États Unis ; aujourd’hui, il y a 80 % d’écart. « Et tout cela avant Trump 2 et avant les conséquences de certaines mesures du, mesures qui vont détruire l’industrie automobile, dévaluer des dizaines de millions de logements, décourager par les excès de normes les initiatives économiques et achever nos agriculteurs, donc appauvrir gravement tout le monde. Au citoyen européen, on dit que sa voiture pollue, que sa maison pollue, que son assiette pollue, que son entreprise pollue ; le sous texte, c’est peut être que sa présence pollue… Ce “plan vert” n’est pas écologiste, il est nihiliste.

« À la mi février, l’Europe devrait présenter, tenez vous bien, un projet de “boussole de la compétitivité”. Il s’agit d’un plan global pour rester dans la compétition mondiale, plan qui devrait annuler ou au moins assouplir un certain nombre de décisions du. Comme dans la bataille entre le nucléaire et le renouvelable – où l’on retrouve d’ailleurs les mêmes camps –, les faits sont en train de donner raison au réalisme et de donner tort aux fanatiques. Mais quel temps, quel argent perdus ! Malheureusement, le climat a peu de choses à voir avec nos règlements kafkaïens. Si l’on prend l’exemple de la voiture, l’effet écologique concret du tout électrique, c’est que l’Europe importera de plus en plus de voitures chinoises, pays qui ne respecte ni l’environnement ni la dignité de ses ouvriers. « La vérité, c’est que nos experts étaient des amateurs, et nos professeurs de vertu des malhonnêtes ! Je vous dis “amateurs”, car ils n’ont pas été capables de réaliser une étude d’impact sur le passage à l’électrique du parc automobile. Une décision aussi grave a été prise avec une légèreté effrayante ! Et je vous dis “malhonnêtes”, parce qu’on a découvert il y a un mois que la Commission européenne avait financé elle même des ONG écolos chargées de faire du lobbying auprès des députés européens. Une telle pratique est évidemment illégale et immorale. Ce que nous dit le fiasco du européen, c’est que ceux qui se présentaient comme le cercle de la raison avaient en fait perdu la raison ; Bruxelles était devenue la nef des fous

tout devient impossible : après la fin de la production de la graine de moutarde française et de la cerise française, nous assisterons peut être à celle de la noisette française, de la pomme française, de la poire française, de la betterave sucrière française… Et la liste pourrait être sans fin

Alors, ouvrons les yeux, arrêtons d’être naïfs et ayons le courage de sortir de l’obscurantisme vert ! Réveillons nous avant qu’il ne soit trop tard pour que la France

nous sommes aujourd’hui réunis dans cet hémicycle pour nos agriculteurs ; pour ceux qui se lèvent chaque matin pour nourrir les Français ; pour ceux qui sont animés par l’amour de leur métier.

En vingt ans, la France est passée du deuxième au sixième rang des exportateurs mondiaux. En vingt ans, nos importations agricoles ont plus que doublé. Notre compétitivité s’effrite excédent commercial agricole est passé de 11,9 milliards d’euros en 2011 à 5,3 milliards d’euros – uniquement grâce aux vins et spiritueux – en 2023. En cinquante ans, nous avons perdu les trois quarts de nos agriculteurs. Les causes du déclin sont nombreuses Les causes du déclin sont nombreuses : surtranspositions mortifères ; avalanches de normes toujours plus contraignantes ; surabondance de réglementations sources de complexité et d’inquiétudes ; injonctions contradictoires en cascade distorsions de concurrence dévastatrices ; politiques publiques court termistes déconnectées des réalités du métier. Nous ne pouvons accepter cette évolution : il est urgent d’agir

Ces diagnostics n’ont pas été suivis d’effets et le mouvement d’érosion s’est accentué. La crise actuelle a même aggravé certaines difficultés et des filières entières sont actuellement menacées, notamment celle de la noisette.

loi a pour ambition première de réarmer la compétitivité de notre agriculture. Il s’agit de permettre aux agriculteurs de trouver des solutions pour développer une production durable

Madame la ministre, l’Europe n’est pas irresponsable ! Une matière n’est autorisée qu’à la condition qu’elle réponde à des critères scientifiques, sanitaires et environnementaux objectifs. Nous devons être plus rationnels

Mes chers collègues, pour enrayer le déclin de notre agriculture, il nous faut affronter les problèmes en face. Voilà ma seule motivation politique

j’ai l’honneur de vous présenter les conclusions des travaux de la commission des affaires économiques relatifs à la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, déposée par nos collègues Laurent Duplomb et Franck Menonville et cosignée par plus de la moitié d’entre nous.

Si la France est une puissance agricole de premier plan, les données sans appel se sont accumulées depuis des années, l’essentiel de nos indicateurs témoigne d’une perte de compétitivité généralisée et, n’ayons pas peur des mots, d’un véritable décrochage de la ferme France. La commission des affaires économiques du Sénat

Les rapports n’ont pas manqué, non plus que les initiatives législatives : une proposition de loi pour la compétitivité de la ferme France a été adoptée ici même en mai 2023. En somme, l’objectif demeure inchangé : redonner de l’air à notre agriculture et la libérer de certaines contraintes, souvent franco françaises, qui non seulement dégradent notre compétitivité

C’est donc au cœur d’une actualité législative déjà forte que nous sommes amenés, mes chers collègues, à nous prononcer sur ce texte. Nous aurions pu croire que le projet de loi d’orientation suffirait, à lui seul, à traiter une bonne partie des questions liées à notre agriculture ; or il n’en est rien.

La tâche n’ayant pas été simple, j’en profite pour saluer l’esprit de responsabilité qui a présidé à nos échanges. Si les auteurs et moi même avons consenti à des compromis, le Gouvernement aussi. Je souhaite remercier une nouvelle fois chaleureusement Mme la ministre de son écoute, de son investissement et de son soutien sur ce texte. Bien sûr, nous ne sommes pas d’accord sur tout – j’y reviendrai –, mais nous avons avancé sur bon nombre de sujets.

à la séparation entre conseil et vente en matière de produits phytopharmaceutiques, qui fait l’objet de l’article 1. Totem pour certains, cette mesure a montré, depuis son adoption en 2018 dans le cadre de la loi Égalim, sa totale inefficacité.

Si je me réjouis que nous soyons parvenus à des compromis sur les deux premiers sujets, je me dois de dire clairement que la question des néonicotinoïdes demeure un point bloquant de nos discussions. L’amendement de suppression déposé par le Gouvernement est, je le dis aussi, inacceptable. Alors que les Premiers ministres et les ministres de l’agriculture se succèdent pour affirmer le principe pas d’interdiction sans solution », ou encore pour annoncer la fin des surtranspositions, nous avons ici une occasion unique de passer de la parole pieuse aux actes concrets. Les filières en situation d’impasse technique

L’article 5 est complémentaire de l’article 15 du projet de loi d’orientation agricole, qui vise à accélérer la prise de décision des juridictions en cas de contentieux, notamment autour de projets d’ouvrages hydrauliques. Il s’agit de déclarer d’intérêt général majeur, sous certaines conditions, les projets de stockage d’eau et les prélèvements qui les accompagnent. a également pour objet d’ajuster la hiérarchie des usages de l’eau, la définition des zones humides ou encore la place de l’agriculture dans les documents de planification de la gestion de l’eau.

Enfin, sur la question des relations entre les agriculteurs et la police de l’environnement, nous avons mené des discussions apaisées pour parvenir à des mesures concrètes susceptibles de permettre de renouer le lien de confiance entre le monde agricole et les inspecteurs de l’environnement.

en l’espace d’un an, notre pays a connu deux mouvements de protestation, dont le premier, d’une ampleur inédite par sa résonance en Europe, a suscité l’émotion de la Nation tout entière. C’est qu’un pays sans paysans n’est qu’un château de cartes. La proposition de loi présentée par messieurs Duplomb et Menonville visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur arrive donc à point nommé.

Je pense tout d’abord à la séparation des activités de vente et de conseil de produits phytopharmaceutiques, qui fait l’objet de critiques de la part et du monde agricole et de rapports parlementaires. Nous voulions plus de conseil

une abrogation totale de toutes les obligations actuelles sans contrepartie n’est pas envisageable. Le Gouvernement propose donc une solution intermédiaire.

Elle est chargée d’évaluer les risques sanitaires et environnementaux posés par des produits phytopharmaceutiques et accomplit ses missions avec précision et responsabilité.

favorable à la pulvérisation par drones, qui permet entre autres de réduire l’utilisation de produits phytosanitaires par une application ciblée. L’expérimentation

Sur la base des modifications introduites en commission, les modalités de consultation ont été considérablement adaptées, ce qui permet de tenir compte de la réalité du projet et de son impact. Pour les projets à plus faible incidence, l’objectif est bien de permettre d’adapter au mieux la procédure et sa charge pour pour l’exploitant. Concernant l’assurance récolte des prairies, la procédure de recours fait l’objet de difficultés constatées sur le terrain, en raison de l’existence d’écarts importants entre le niveau de pertes issues de l’indice et celui qui est constaté empiriquement par l’éleveur. Pour autant, il n’est ni possible ni souhaitable de revenir à un système d’expertise de terrain basé sur des bilans fourragers et sur une reconnaissance collective des pertes, à l’instar du régime précédent des calamités agricoles, que la loi a réformé. Cela acterait la fin de l’assurance prairie en raison du retrait immédiat des assureurs et des réassureurs de ce segment de marché, pour lequel une expertise de terrain est incompatible avec une évaluation indicielle des pertes.

de renforcement de l’offre d’assurance récolte destinée aux prairies. Il s’agit d’accompagner son développement et d’assurer son appropriation par l’ensemble des acteurs. Je sais que des échanges sont en cours entre les sénateurs, les assureurs et les professionnels pour améliorer le système. Le Gouvernement est prêt à prendre sa part

nous nous sommes saisis. Ainsi, en lien avec le ministère de la transition écologique, nous avons proposé une rédaction permettant de répondre aux enjeux soulevés. Sans revenir sur la définition,

nous créons une catégorie de « zones humides fortement modifiées », par analogie avec la catégorie de « masses d’eau fortement modifiées », prévue par la directive cadre sur l’eau.

jours tout comme je condamne les propos malheureux qui n’ont fait que jeter de l’huile sur le feu. C’est justement pour mettre fin à ces crispations que nous poursuivons les travaux engagés en vue de privilégier les contrôles administratifs par rapport aux contrôles judiciaires et, plus globalement, de limiter les contrôles. Pour cela, il est important de coordonner l’ensemble des services l’État. C’est le sens de la création des missions interservices agricoles (Misa), pilotées par les préfets de département, en appui des missions interservices de l’eau et de

Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, la position du Gouvernement sur ce texte. J’ai essayé d’être la plus précise possible, car je sais le travail très important que vous avez fourni pour lui permettre d’aboutir. Les objectifs que nous cherchons à atteindre sont les mêmes. Je me réjouis donc

Les nombreuses régressions que contient cette proposition de loi sont un condensé des démarches et pratiques les plus néfastes défendues par l’agro industrie. Revenons quelques années en arrière. Il y a vingt ans, le Parlement, réuni en Congrès, votait à l’unanimité la Charte de l’environnement. Notre pays se plaçait ainsi en précurseur de la protection du vivant et de la biodiversité. Ce texte, comme vous le savez, a intégré le bloc de constitutionnalité lors de la révision constitutionnelle du 1 mars 2005.

en discussion ne définit aucun cadre légal suffisant pour protéger le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, pourtant garanti par l’article 1 de la Charte de l’environnement. Cette proposition de loi est également une attaque en règle contre le droit européen.

Les dispositions du présent texte, contraires au droit européen, exposent clairement la France à des amendes. L’argent public serait mieux investi dans des dispositifs visant à accompagner la transition agroécologique Dans sa décision du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a consacré la préservation de l’environnement comme enjeu supérieur à la liberté d’entreprendre. ainsi reconnu que « la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle » pouvant justifier des atteintes à la liberté d’entreprendre. Par une décision du 10 décembre 2020, le Conseil constitutionnel a précisé que les limites apportées par le législateur à l’exercice du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, consacré par l’article 1 de la Charte de l’environnement, « ne sauraient être que liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi.

à un motif d’intérêt général. Lever l’interdiction des remises, rabais et ristournes à l’occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques est contraire à l’avis du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), qui recommande d’éviter toute incitation commerciale pouvant conduire à l’utilisation inappropriée des pesticides. J’en viens à l’épandage par drones, à l’article 2. La loi Égalim prévoyait la mise en place d’une expérimentation relative à la pulvérisation aérienne de précision de produits phytopharmaceutiques,

Par ailleurs, dans un arrêt du 12 avril 2013, le Conseil d’État a jugé que l’existence d’un tel risque devait être regardée comme une « hypothèse suffisamment plausible en l’état des connaissances scientifiques pour justifier l’application du principe de précaution

une nouvelle définition des zones humides, ce qui amoindrit leur protection, la reconnaissance d’un caractère d’intérêt général majeur pour les mégabassines ou encore la nouvelle réglementation que vous souhaitez appliquer aux ICPE. Le rapporteur a d’ailleurs réduit à peau de chagrin la consultation du public, déjà fortement affaiblie par loi Industrie verte, pour tous les projets soumis à autorisation environnementale, pas seulement pour les ICPE agricoles.

doutons fortement de la compatibilité du texte avec la directive cadre sur l’eau, notamment en ce qui concerne le respect des objectifs de reconquête du bon état écologique des masses d’eau.

Alors que les sécheresses, les preuves de l’impact des pesticides et la pollution de notre ressource en eau devraient nous pousser à accélérer la transition, on voudrait nous contraindre à ralentir. Pire, on nous propose même de faire marche arrière en revenant sur les trop rares avancées acquises ces dernières années. Par ailleurs, il est crucial de mettre fin à cette opposition factice entre économie et environnement. Cessez d’opposer agriculteurs et écologistes, car notre destinée est commune. Les normes environnementales permettent de protéger la santé des agriculteurs et les services écosystémiques indispensables rendus par la biodiversité. S’attaquer à ces normes, c’est s’attaquer à la durabilité de l’agriculture française.

dans l’enceinte de cet hémicycle que nous devons peser chacun des enjeux, confronter les idées et, si possible, proposer des solutions équilibrées. En tout cas, c’est en ce sens que j’ai travaillé avec le Sénat.

Ce débat est d’autant plus important que l’agriculture est un secteur fondamental, vital à la fois pour notre économie, pour nos territoires et pour notre sécurité alimentaire.

pour l’écosystème, le présent texte prévoit de lever les quelques protections qui ont été intégrées de haute lutte dans notre code de l’environnement. La réautorisation des néonicotinoïdes, la pulvérisation aérienne de pesticides, la mise en danger des zones humides et la fragilisation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de

opposé à cette nouvelle manœuvre dilatoire, alors que l’agriculture requiert toute l’attention du politique. L’agriculture doit être soutenue pour accomplir une transition qui se veut agroécologique.

à ne pas vouloir regarder la réalité en face ! Continuez à mettre les agriculteurs dans un corner ! Continuez à faire croire qu’une solution miracle est possible. La seule chose que vous récolterez, c’est que les agriculteurs ne seront plus agriculteurs et que les paysages ne seront plus ceux

Et maintenant que les fermes ont disparu, que ce sont toujours les plus petits qui se cassent la gueule, qui disparaissent ou se suicident, vous mettez sur le dos des écologistes

Nous allons aborder des sujets délicats et nous aurons des désaccords. Toutefois, je crois fondamental de montrer, une fois encore, que le Sénat est un lieu de réflexion sérieux et utile pour la France.

Comme s’il n’était pas assez exposé aux aléas du climat, force est de constater que nous y avons collectivement ajouté des contraintes normatives parfois inutiles, quelques fois invivables. Certaines sont justifiées, mais la nécessité de simplifier s’impose à nous. Nous l’avons entendu à chaque manifestation et à chaque rassemblement des professionnels depuis maintenant plus d’un an : nos agriculteurs veulent être écoutés et, surtout, voir les promesses se traduire en actes. de cette proposition de loi vont dans le sens d’une simplification. Je pense ainsi à l’article 3, qui concerne la simplification du régime français des installations classées pour la protection de l’environnement. L’allégement de la procédure sera bien évidemment salué par les professionnels.

Pourtant, face aux sécheresses et aux déséquilibres de la pluviométrie, nous devons agir pour déclarer les ouvrages ayant vocation à prélever et stocker de l’eau à des fins agricoles comme étant d’intérêt général majeur. ci sont en effet particulièrement nécessaires pour nos agriculteurs, qui souhaitent garder une agriculture de qualité malgré les effets du dérèglement climatique.

Selon Météo France, 2024 figure parmi les dix années les plus marquées par la pluie depuis 1959 à l’échelle nationale, avec une pluviométrie de plus de 15 % au dessus de la moyenne. N’oublions pas non plus les efforts de sobriété que nous pouvons toutes et tous réaliser afin d’éviter tout gaspillage.

d’éviter autant que faire se peut des procédures judiciaires dès lors que les faits poursuivis relèvent d’une primo infraction ou d’une infraction ayant causé un faible préjudice environnemental.

il a bien été précisé en commission que le ministre devra statuer selon les mêmes critères que ceux du directeur général de l’Anses, qui relèvent du droit européen. De plus, le ministre de l’agriculture pourra demander à l’Anses d’examiner par priorité un dossier en matière phytopharmaceutique, afin de mieux répondre aux demandes urgentes émanant de filières se trouvant dans une impasse technique. Je crois que ces mesures sont attendues par les agriculteurs. Nous devons en effet stopper les surtranspositions du droit européen dans le droit français et appliquer le principe « pas d’interdiction sans solution » à nos politiques agricoles.

Je vous remercie,

au tout ou rien, préférons la nuance. Ce texte de nos collègues Duplomb et Menonville a le mérite de cerner un enjeu : l’évolution du métier d’agriculteur et de ses contraintes. Je comprends pleinement son fondement, à l’instar de la profession. Nos paysans s’élèvent contre la surtransposition, les accords commerciaux internationaux et la lourdeur administrative, notamment française. À quelques semaines des élections des chambres d’agriculture, les syndicats se sont mobilisés pour faire entendre la souffrance des femmes et des hommes de la terre. En colère contre le Mercosur, étranglés par des trésoreries exsangues après des années frappées par de mauvaises récoltes et des aléas climatiques, sanitaires et économiques, leurs attentes sont fortes.

mon père avait des tracteurs et des produits de synthèse ; je suis passé à la machine à vendanger et j’ai converti mon exploitation au bio ; enfin, mon fils gère le domaine avec une tablette et utilisera à coup sûr des robots…

? Celui de la dépendance envers l’industrie, sans oublier le coût écologique et de santé publique dont nous n’avions pas conscience avec l’éradication, par exemple, de beaucoup d’insectes et d’oiseaux, l’appauvrissement des sols en matière organique et l’apparition de maladies souvent mortelles pour nos agriculteurs. De l’histoire, puisons le bon. L’agriculture a su évoluer, avec la haute valeur environnementale et les agricultures raisonnée et bio, aux côtés d’une agriculture conventionnelle, qui s’est adaptée aux objectifs environnementaux. Nous pouvons atteindre une agriculture plurielle répondant aux différents enjeux économiques, environnementaux et de santé publique, qui doivent rester équilibrés. Pourquoi opposer des modèles ? Pourquoi s’imposer des œillères ?

Pour les néonicotinoïdes, n’ayons pas peur du débat. Ils ne doivent pas être le sujet qui fâche : nous pourrions nous entendre sur des interdictions ciblées, lorsque les produits de substitution n’existent pas.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui une proposition de loi importante pour l’avenir de notre agriculture, un secteur que nous savons en crise et confronté à des défis historiques. Les réglementations françaises, souvent excessivement contraignantes et parfois mal adaptées à la réalité du terrain, aggravent ces difficultés. Ce texte ne doit rien au hasard : il s’inscrit dans le contexte particulier d’une agriculture en souffrance et résulte de nombreux travaux menés par le Sénat au cours des dernières années. Dès 2022, la commission des affaires économiques alertait sur la perte de compétitivité de notre agriculture par rapport à nos voisins européens. Les surtranspositions et la surréglementation françaises sont alors identifiées parmi les freins au développement de nos filières agricoles. Cette situation préoccupante s’est aggravée au fil du temps, comme en témoigne la diminution de l’excédent commercial alimentaire de la d’euros à 5,3 milliards entre 2011 et 2023. Nos agriculteurs, souvent épuisés par la charge administrative, ont encore à subir des normes lourdes et inadaptées. C’est dans ce contexte que le mouvement de contestation a émergé, début 2024.

de simplifier les démarches administratives et de restaurer la compétitivité de notre agriculture. La proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France, adoptée en 2023, qui tend à lever de premiers obstacles réglementaires, y contribue.

pour objet de faciliter la gestion de la ressource en eau, répond également à une nécessité. L’agriculture doit bénéficier de l’irrigation sans être freinée par une législation déconnectée des réalités du terrain. La France ne peut se permettre une incertitude sur la gestion de l’eau, que les agriculteurs considèrent comme la plus précieuse des ressources. Ainsi, cette proposition de loi est le fruit de plusieurs années de réflexion. Elle regroupe un ensemble de propositions concrètes tendant à lever les entraves agricoles, améliorer la compétitivité de la ferme France et répondre à des besoins urgents. chers collègues, cette proposition de loi est une évolution, non une révolution. Elle vise à lever des obstacles bien identifiés et à redonner des marges de manœuvre à nos agriculteurs, afin qu’ils puissent rivaliser sur un pied d’égalité avec leurs voisins européens et mondiaux.

s’il est vrai que l’agriculture ne fait pas toute la ruralité, il n’est pas moins vrai qu’il n’y a pas de ruralité vivante sans agriculteurs. Dès lors, l’agriculture représente un double enjeu

l’on peut discuter et critiquer les excès de paperasserie et de bureaucratie, on peut assurément simplifier sans aggraver les précarités et les insécurités ni sacrifier la vie sur notre planète.

sur les fourches à fumier des tracteurs, des mots d’ordre contre les normes. Dans un gigantesque tête à queue confusionniste,

et même aux locaux départementaux de la Mutualité sociale agricole (MSA), qui est pourtant la sécurité sociale des paysans. Dans le département des Côtes d’Armor, nous avons la fierté d’accueillir un grand campus de recherche regroupe, sur le Zoopôle de Saint Brieuc Ploufragan, près de 1 000 chercheurs et scientifiques, ce qui en fait vraisemblablement

Ces laboratoires produisent des études, mettent au point des vaccins, formulent des préconisations de méthode… Ils ne sont donc pas un problème pour notre agriculture ; au contraire, ils trouvent généralement des solutions aux problèmes et pathologies multiples

Nous avons ainsi besoin d’une autorité scientifique indépendante, apte à objectiver les situations et à apprécier les risques et habilitée à homologuer les produits.

à effacer toutes les normes et préconisations… Cette proposition de loi est, à nos yeux, un retour au passé. Elle ne réglera pas le problème du cheptel breton, qui a perdu 120 vaches par jour au cours de l’année écoulée.

Au recours à la tronçonneuse, nous préférons le bien commun, parce qu’il y va aussi de la survie de l’humanité. Telles sont les raisons qui nous conduisent à nous opposer à cette proposition

les exploitations grossissent au détriment de la vitalité de nos communes rurales ; notre agriculture souffre d’une incapacité à s’adapter et se protéger face aux changements climatiques et aux crises sanitaires qui se succèdent, et j’en passe ! En quelques décennies, nous avons rendu notre agriculture paysanne et locale dépendante dépendante d’autres puissances, des marchés financiers, de la crise énergétique. De perte de repères en perte de sens, nous nous sommes perdus. Tel est le bilan de soixante dix ans de politique agricole au service de la productivité coûte que coûte, que coûte, de l’agrobusiness, des firmes agrochimiques, des banques, des spéculateurs, mais certainement pas au service des paysans, de la terre, de l’eau et de ce qui nous fait vivre. Tel est le bilan d’orientations dictées depuis toutes ces années par le syndicat majoritaire, plus attaché à développer les biocarburants et l’exportation bas de gamme qu’à répondre au mal être et à la détresse des agriculteurs.

Permettez moi de vous dire, chers collègues Duplomb et Menonville, qu’avec ce texte caricatural, loin du bon sens paysan, vous vous transformez en docteurs Folamour de l’agriculture.

Hier, vous vous attaquiez à 61 200 fermes en bio, pour 2,76 millions d’hectares, en proposant, et en obtenant, avec l’aval de la ministre, la suppression de l’Agence Encore un contresens et une insulte à des milliers de paysans ; même la FNSEA ne vous suit pas sur ce chemin. Considérez vous vraiment que c’est rendre service aux agriculteurs que de réautoriser les promotions sur les pesticides et d’affaiblir l’Anses ? Combien de temps allez vous faire perdurer ce mensonge sur la dangerosité des pesticides ? Combien de temps assumerez vous d’exposer les agriculteurs aux cancers de la prostate, à Parkinson, à l’infertilité et à d’innombrables maladies ? Le fonds d’indemnisation des victimes des pesticides traite plusieurs centaines de dossiers par an. Ces images terribles d’agriculteurs découvrant chez le médecin que leur métier les empoisonne ne nous touchent elles donc pas ? Mes chers collègues, pourquoi vous en prendre à ce point aux apiculteurs en réautorisant des néonicotinoïdes – trois substances, et non une seule, comme je l’ai entendu. L’Union nationale de l’apiculture française (Unaf) vous interpelle directement

à l’agriculture représente jusqu’à 5 milliards d’euros pour les seuls services de pollinisation. Mes chers collègues, pensez vous sincèrement qu’en autorisant l’épandage par drone, vous rendez service aux agriculteurs ? Pensez vous les aider en aggravant leur dépendance à des technologies onéreuses à l’efficacité non démontrée et en creusant leur endettement ? Mes chers collègues, pensez vous vraiment aider les paysans en favorisant l’effondrement de la biodiversité, l’empoisonnement et l’accaparement de l’eau ? Dans un monde où l’eau potable se raréfie, où les sécheresses se multiplient, considérez vous sérieusement que nous devons, que nous pouvons, continuer à la gaspiller davantage ? Madame la ministre, à quoi va donc servir la conférence sur l’eau promise par le Premier ministre si cette proposition de loi confiscatoire est adoptée dans cette rédaction ? Mes chers collègues, pensez vous aider les paysans en détruisant toute la démocratie environnementale et ce qu’il reste de concertation et de consultation du public, préalable à l’installation de la plupart des activités économiques qui emportent inévitablement des conséquences sur nos territoires et sur nos lieux de vie ? nos lieux de vie ? Il est encore temps de faire appel à votre bon sens paysan, à celui qui écoute la nature, son évolution, qui sait s’adapter, ce bon sens qui a permis à l’agriculture de traverser des millénaires en conservant une terre fertile, que nous venons de mettre à mal en quelques décennies. Il est encore temps de renouer avec la logique de René Dumont, qui disait : « Regardez bien votre vache, c’est un animal extraordinaire ; elle a une barre de coupe à l’avant, et un épandeur à l’arrière. Si vous flanquez cet animal dans le milieu d’un pré, elle fait le travail toute seule. » Mes chers collègues, revenez au bon sens !

ne parviennent pas à vivre de leur travail ; oui, la mondialisation déloyale fragilise plusieurs de nos filières ; mais non, la bonne réponse au malaise agricole n’est pas l’assouplissement des règles encadrant l’usage des pesticides, non

À l’heure de nous prononcer sur ce texte, remémorons nous les termes de la Charte de l’environnement de 2004. Son préambule dispose que « les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ».

au malaise du monde agricole. Comment expliquer que, en France, puissance agricole historique, capable pendant des siècles de nourrir une population toujours croissante par ses propres ressources, des centaines d’agriculteurs mettent fin à leurs jours chaque année ? Comment tolérer que des contraintes administratives absurdes, des importations dérégulées et des normes excessives menacent aujourd’hui la pérennité même de notre agriculture ? ? Pourtant, tandis que l’on accable nos agriculteurs de surtranspositions et de réglementations disproportionnées, les responsables politiques n’hésitent pas à signer en toute discrétion des traités comme l’accord

Néanmoins, ce que la politique a défait, nous avons ici le pouvoir de le refaire. Les attentes de nos agriculteurs sont simples et légitimes : vivre dignement de leur travail, être protégés d’une concurrence internationale déloyale et voir lever les lourdeurs bureaucratiques qui entravent leur activité. Faciliter la vie de nos agriculteurs, tel est le mérite de cette proposition de loi. Par exemple, nous approuvons l’article 1, qui abroge l’interdiction en France des remises, rabais et ristournes sur les produits phytosanitaires, alors que les Espagnols ou les Allemands, nos premiers concurrents, peuvent négocier le prix de leurs produits.

Entre l’urgence économique du monde agricole et l’inquiétude écologique d’une partie de nos concitoyens, il est à l’honneur des auteurs de ce texte d’avoir su nous soumettre une rédaction équilibrée. Cette proposition de loi constitue une première étape. Il faut mettre fin à toutes les surtranspositions de normes européennes, réduire les charges administratives et fiscales inutiles et garantir des revenus dignes à ceux qui travaillent sans relâche pour nourrir nos concitoyens. Ce sera tout l’objet du projet de loi d’orientation agricole, dont le Sénat se saisira dans les prochaines semaines. Néanmoins, nous devons également financer la recherche de solutions pour assurer la vigilance sanitaire nécessaire à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et aboutir, à terme, à une production sûre pour nos agriculteurs, tout en protégeant la santé publique et l’environnement.

Merci,

nourrit l’excellence de nos filières agroalimentaires, mais les boulets sont trop nombreux et sapent leur compétitivité. Les politiques climatiques engagées par l’Union européenne sont légitimes et ambitieuses au regard des enjeux, mais elles ne doivent pas induire une séparation entre les producteurs et les 450 millions de consommateurs. La confiance dans l’alimentation reste capitale pour nos agriculteurs. Nombreux sont ceux qui veulent laver plus blanc que blanc et la France, cherchant sûrement à bien faire, a très largement surtransposé les directives européennes. Les parlementaires et la représentation nationale l’ont fait avec la certitude que nos partenaires européens partageaient cette croyance. Surtransposition, interdiction arbitraire de produits phytosanitaires, définition trop contraignante des zones humides, impossibilité de préserver la ressource en eau : nous ne pouvons plus laisser autant de distorsions de concurrence à l’intérieur même de l’espace européen qui, je le rappelle, est la zone la plus écologique du monde. Alors, mes chers collègues, je remercie publiquement les sénateurs Duplomb et Menonville. Oui, vraiment, sincèrement : merci ! Cette proposition de loi est la première et la seule à répondre aux attentes des agriculteurs et des producteurs français. français. Je vous le dis le plus sérieusement du monde : oui, tous les agriculteurs français sont convaincus par la nécessité d’effectuer des efforts sur les enjeux écologiques. Ils sont attachés, ancrés à leur sol, à leur territoire, à la nature environnante : ils y vivent. C’est bien pour cela que l’agriculture européenne est la plus saine, la plus sûre et la plus respectueuse du bien être animal de la planète. Nous avons déjà baissé de 95 % l’utilisation des pesticides cancérogènes, mutagènes et l’administration d’antibiotiques dans nos élevages. Mais on ne peut pas tout supprimer si l’on veut lutter contre les maladies animales. Dans le même temps, nous subissons une augmentation massive des importations de produits agricoles ne répondant pas aux mêmes contraintes de production : 60 % pour les fruits, 40 % pour les légumes. Je ne vous parle même pas de l’emblème des importations : le

stagner et nous ne pourrons plus enrayer la chute. Notre balance commerciale de produits agricoles, excédentaire de 5 milliards d’euros, s’est déjà repliée de 43 %. Depuis plus d’un an, les agriculteurs manifestent, en souffrance depuis bien plus longtemps encore et nous disent systématiquement : « Laissez nous faire notre travail, notre métier, et bien vous nourrir durablement avec des produits sains et de qualité.

Comme Rome, l’agriculture de demain ne se fera pas en un jour. Tout le monde est prêt à applaudir les grandes déclarations en vue de changer les choses entendues lors des crises, mais, hélas ! nous attendons encore les actes. Les agriculteurs patientent, nous leur avons fait beaucoup de promesses, nous avons suscité beaucoup d’espoirs, mais depuis un an,

agricole, bien qu’incomplet, est toujours en discussion ; les simplifications promises par le Gouvernement Attal attendent que l’administration accepte enfin de réduire le réglementaire et de pondre arrêtés et décrets. nous ne produisons que du rien et, à cause de cela, l’agriculture part dans le décor. Notre ambition paraît tellement légitime, tellement simple à mettre en œuvre, et pourtant, le constat est terrible : les gouvernements sont tétanisés par la peur des attentes sociétales, par la peur des sondages. Seulement voilà, tout le monde est coincé dans une temporalité qui nous échappe. Le salon de l’agriculture arrive et la mauvaise volonté va finir par se Pour nous, parlementaires, elle est déjà bien visible : pas de marche arrière, vous crantez la ceinture qui étrangle l’agriculture, et cela commence à se voir.

besoin. Pendant les débats, je serai sans concession avec les marchands de peur et avec les administrations, d’autant que certaines d’entre elles nous ont caché des éléments pendant les auditions. Madame la ministre, je sais que je peux vous faire confiance, mais je vous demanderai tout de même quelques explications et j’attendrai des réponses. Les agriculteurs savent que nous leur mentons, il est temps d’arrêter d’avoir peur, peur des drones, peur des nouvelles techniques génomiques, peur de stocker l’eau. Nous avons peur de notre ombre ! Nous sommes devenus des Gaulois effrayés que le ciel ne leur tombe sur la tête. Or nos ambitions doivent être immenses pour que nous restions dans la course des grands équilibres mondiaux. Je vous le demande avec force, mes chers collègues : soyons courageux, gardons un cap ambitieux face aux changements climatiques, mais rectifions les excès.

Face à ces constats, il est impératif de redonner de l’air à nos agriculteurs pour leur permettre de vivre dignement de leur travail, de produire et de garantir la souveraineté alimentaire de notre pays. Le secteur de l’élevage est particulièrement touché, confronté à l’apparition de nouvelles épizooties qui emportent des conséquences sur l’ensemble de la chaîne ; il souffre tout autant des procédures environnementales complexes et coûteuses. Or il est un pilier essentiel de notre agriculture et recèle un savoir faire important en France. Au cœur de l’économie agroalimentaire, de ses filières et des divers emplois qu’elles induisent, il est le poumon de nos campagnes. nos campagnes. Il assure une production de qualité et un approvisionnement local, il contribue à l’entretien de l’espace, au maintien de l’ouverture des paysages et à la préservation de la biodiversité. Laisser l’élevage français s’effondrer serait renoncer à une part de notre identité, de notre patrimoine et de notre avenir. La simplification est une nécessité pour ne pas désespérer des acteurs qui savent faire preuve de bon sens et qui ont déjà bien assez de

et permettra de libérer l’activité agricole de normes lourdes et contradictoires. Elle est aussi complémentaire du projet de loi d’orientation agricole que nous allons examiner dans les prochaines semaines ont pour objectif de consolider la souveraineté alimentaire et agricole de la France en affichant une ambition programmatique, tout en apportant des réponses immédiates pour promouvoir une agriculture compétitive et durable.

Sur ces quatre sujets, cette proposition de loi apporte des solutions. Elle met fin aux normes françaises excessives qui pénalisent certaines filières par rapport à leurs concurrents européens.

garantit un accès sécurisé à l’eau pour l’agriculture avec l’inscription dans la loi d’un principe de non régression du potentiel agricole par la politique de l’eau. Il s’agit de prendre en compte la place de l’usage agricole dans la hiérarchie des usages de la ressource et de traiter les projets de stockage d’eau à usage partagé, facilitant ainsi la mise en place de solutions visant à améliorer l’accès à l’eau pour l’agriculture. Enfin, elle promeut une relation plus apaisée avec les services de contrôle par un dialogue et des solutions amiables. Ce texte apporte des évolutions nécessaires et a le mérite de traiter les sujets qui concernent l’activité quotidienne des agriculteurs, d’améliorer la « vivabilité » ressentie par les agriculteurs. En conclusion, ce texte contribue, à mes yeux, à améliorer notre modèle de souveraineté agricole et à soutenir une agriculture compétitive, durable et économiquement viable, présente sur tout le territoire, montagnes, plaines, vallées, bref, en milieu rural.

je tiens tout d’abord à saluer mes collègues Laurent Duplomb et Franck Menonville pour cette proposition de loi qui revient sur un certain nombre de dispositifs législatifs que nous savons aujourd’hui préjudiciables à notre économie rurale et à notre souveraineté agricole. Je le dis d’autant plus aisément que j’ai été rapporteur de l’ensemble des lois Égalim depuis 2018.

Ce texte vient répondre aux dysfonctionnements et aux incohérences pointés par les agriculteurs afin de rendre à l’agriculture française des marges de compétitivité au nom de la souveraineté alimentaire.

Face à ces impasses techniques, l’interdiction met en difficulté les producteurs français de betterave, ce qui explique la dérogation encadrée de 2020 et 2023. Les producteurs de noisettes, de pommes de terre et bien d’autres se trouvent également en grande difficulté,

La survie de notre agriculture, sa compétitivité au regard de ses concurrents à la fois internationaux et européens, le principe de « non interdiction sans solution » sont autant de motifs qui doivent nous amener à desserrer les contraintes franco françaises pesant sur nos agriculteurs. En ce sens, notre groupe proposera, sur l’initiative d’Anne Sophie Romagny, deux amendements sur le modèle de ce qui a été fait pour les betteraves, afin de rassurer sur cette mesure, d’encadrer l’usage et, enfin, de s’aligner sur la réglementation européenne. De la même manière, la séparation entre vente et conseil ainsi que l’obligation d’un conseil stratégique indépendant n’ont pas conduit à une diminution des volumes de produits utilisés en France. Il est donc légitime de revenir sur ces dispositions qui engendrent des surcoûts, alors que le préconisera un diagnostic modulaire qui permettra de mieux évaluer la viabilité économique et écologique d’une exploitation agricole. La proposition de loi revient également sur l’usage des drones, lequel n’est pas remis en cause par l’Anses. Je présenterai pour ma part un amendement visant à mieux répondre aux difficultés auxquelles sont confrontés nos viticulteurs.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous étudions aujourd’hui ne me paraît pas contenir de solutions pertinentes pour la défense de notre agriculture et de nos agriculteurs.

Il faut assurer des prix rémunérateurs en mettant en place un véritable encadrement des marges dans la chaîne de valeur afin de garantir des prix équitables, de lutter contre les abus de certains intermédiaires et d’encourager les circuits courts et locaux, bien que ces derniers – j’en suis conscient – ne soient pas la solution unique. Il faut également alléger les démarches administratives et rendre les contrôles

il est souhaitable d’investir massivement dans des filières biologiques et de qualité pour capter de nouveaux marchés. Le récent vote du Sénat supprimant l’Agence bio va totalement à rebours de ce qu’il faut faire et provoque, à raison, l’incompréhension des acteurs de la filière. Ce n’est pas en affaiblissant ou en supprimant des structures de recherche que nous rendrons service à notre agriculture. L’utilisation de produits dangereux affecte en premier lieu la santé des agriculteurs eux mêmes. C’est pourquoi je m’oppose à l’article 2 de la présente proposition de loi, qui remet en cause le cadre existant en matière d’autorisation et d’usage des pesticides. Il affaiblit la position de l’Anses tout en revenant sur des interdictions actées.

Ces évolutions se feront grâce à la science, grâce aux recherches menées par les différents organismes qui accompagnent nos agriculteurs et par les agences dont les auteurs de la présente proposition de loi veulent démagogiquement limiter l’influence. Ce n’est pas en cassant le thermomètre que l’on fait baisser la température Il est un combat primordial, celui que la France doit mener également au niveau européen, afin de garantir que les produits agricoles importés respectent les mêmes normes environnementales, sanitaires et sociales que celles qui sont imposées aux agriculteurs français. La France doit être intraitable : tout produit ne respectant pas nos règles sanitaires et sociales ne doit pas être commercialisé en France. C’est ce que l’on appelle les clauses miroirs. Je suis convaincu que les recettes que contient cette proposition de loi ne permettront pas d’améliorer la situation de nos agriculteurs. La dérégulation, le libéralisme économique à tout va sont, au contraire, à l’origine des difficultés que traverse l’agriculture française depuis des années.

c’est avec une profonde conviction et un sentiment d’urgence que je prends aujourd’hui la parole pour soutenir la proposition de loi de nos collègues Laurent Duplomb et Franck Menonville, un texte essentiel qui vise à répondre aux défis critiques auxquels est confrontée l’agriculture de notre Cette proposition de loi emporte un engagement fort en faveur de nos agriculteurs, de nos territoires et, au delà, de la souveraineté alimentaire de notre pays. pays. En Lot et Garonne, département agricole par excellence, cette crise est particulièrement perceptible. Les exploitants spécialisés dans les fruits, les légumes ou l’élevage

Confrontés à une urgence phytosanitaire liée à des ravageurs, nos producteurs se retrouvent dans une impasse absurde du fait de l’interdiction en France de l’acétamipride, un produit pourtant autorisé dans d’autres pays européens.

permettrait de garantir à nos agriculteurs qu’ils disposeront des outils nécessaires pour préserver leur production et faire face à des situations exceptionnelles.

En laissant entrer sur notre marché des produits issus de pratiques agricoles interdites en France, nous exposons nos agriculteurs à une concurrence déloyale.

L’un des leviers clés de cette souveraineté est la gestion de l’eau, un enjeu crucial dans un contexte de changement climatique. Aujourd’hui, trop de projets de retenue d’eau et de lac collinaire sont retardés ou bloqués par une administration lourde et complexe.

de sécuriser l’irrigation, de pérenniser les exploitations agricoles et de préparer notre pays aux défis climatiques à venir. Le modèle agricole français repose sur trois piliers essentiels : la diversité des productions, la qualité des produits et le lien étroit avec le territoire, car nos agriculteurs façonnent nos paysages, maintiennent la vie rurale et préservent nos traditions.

En soutenant cette proposition de loi, nous affirmons que la France protège ses agriculteurs et ses filières stratégiques, que la concurrence internationale doit être équitable et reposer sur des normes communes respectées par tous, que la souveraineté alimentaire de la France n’est pas négociable. En adoptant ce texte, nous envoyons un signal clair à nos agriculteurs : nous avons entendu leur appel.

contre 400 000 aujourd’hui. Près d’un quart des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté, un taux bien plus élevé que dans toutes les autres catégories socioprofessionnelles. Un agriculteur sur cinq ne parvient pas à dégager un revenu suffisant pour se rémunérer à la fin du mois. Et chaque année, ce sont près de 300 agriculteurs qui se suicident de désarroi. Derrière ces chiffres, derrière ces statistiques parfois tragiques, il y a des femmes et des hommes, ces héros de nos territoires, véritables piliers de nos communes, qui se trouvent confrontés à des contraintes de plus en plus lourdes qui entravent leur capacité à exercer le métier le plus noble du monde. Il est de notre devoir, au Sénat, de leur apporter les réponses qu’ils attendent. Défendre nos agriculteurs, c’est d’abord reconnaître la complexité de leur quotidien. Ils sont soumis à des normes, notamment européennes, qui, bien que parfois inspirées par de bonnes intentions, ne tiennent pas compte des réalités.

Combien de fois avons nous entendu des exploitants se plaindre de passer plus de temps derrière leur bureau qu’à travailler dans leur champ ou dans leur étable ? Ces heures perdues sont des heures volées à leur passion, à leur production et, finalement, à notre souveraineté alimentaire. Il est de notre responsabilité de réaffirmer la place stratégique de l’agriculture dans notre pays, Face à la concurrence européenne, parfois déloyale, face aux crises économiques et climatiques, nous devons offrir à nos agriculteurs des outils pour rester compétitifs. rester compétitifs. Défendre nos agriculteurs, c’est enfin défendre nos territoires ruraux, nos paysages et notre patrimoine. Chaque exploitation qui disparaît, c’est une parcelle de France qui s’éteint. Nous ne pouvons pas accepter ce déclin silencieux, car lorsque la flamme de l’agriculture vacille, c’est une part de l’âme française qui risque l’extinction. Mes chers collègues, en votant ce texte, après des débats sans nourris, nous affirmerons notre soutien à celles et à ceux qui travaillent sans relâche pour garantir notre souveraineté alimentaire. Nous leur montrerons que la République est à leur côté. Il est grand temps d’alléger le fardeau de nos agriculteurs et de leur redonner les moyens de réussir.

Arrêter tout contrôle sur les pesticides épandus sur nos sols ? Déverser des pesticides sur nos sols jusqu’à l’épuisement des stocks et des sols ? Faire croire à nos exploitants qu’il n’y aura plus de contrôle du tout

du point de vue de l’usage des produits phytosanitaires ne peut précisément être évalué, mais les auditions conduites par vos rapporteurs laissent penser qu’il est faible, notamment en raison des effets contre productifs que la réforme a pu produire, mais aussi de sa faible application. » Ils ajoutent que « le passage d’un conseil formalisé formulé par les vendeurs à une absence de conseil ou à un conseil oral et informel paraît avoir diminué la qualité du conseil délivré et laissé un certain nombre d’agriculteurs “orphelins”

On tente, on essaie avec de bonnes intentions, mais si l’on s’est trompé dans les modalités de réalisation d’un objectif, il faut le reconnaître et le faire évoluer.

pour prévenir les conflits d’intérêts. Ensuite, l’activité de conseil restera interdite aux fabricants de produits phytopharmaceutiques pour éviter précisément tout conflit d’intérêts.

le prosulfocarbe est un pesticide qui est utilisé sur les céréales et qui a contaminé de nombreux lots d’agriculteurs biologiques.

Cette interdiction, qui existe dans d’autres domaines tels que la vente de médicaments vétérinaires, a montré son efficacité pour limiter l’importance de l’argument commercial dans le choix des produits par le décideur. donc lieu de privilégier le conseil plus que la ristourne et d’écarter les risques d’interférence avec des considérations commerciales. Je rappelle que cette interdiction, telle qu’elle figure actuellement dans le code rural et de la pêche maritime, ne porte pas sur les produits de biocontrôle. Elle ne s’oppose donc pas à l’essor de ces produits que le Gouvernement cherche à promouvoir.

et ont suffisamment de discernement pour acheter au bon moment et de la bonne manière. Sur le plan de l’efficacité,

évoquée, nous consentirons à maintenir cette interdiction et nous donnerons donc un avis favorable.

toutes les structures qui s’intéressent au bio, et elles sont très nombreuses. La question qui se pose est de savoir comment favoriser une meilleure synergie

un malentendu dont je dirais qu’il a été largement entretenu, il n’est pas question de diminuer l’appui budgétaire, financier ou structurel que le Gouvernement, et singulièrement mon ministère, entend apporter à l’agriculture biologique, que j’ai toujours défendue à titre personnel, et cela depuis très longtemps. Je crois que l’agriculture biologique

l’on est attaché, comme vous le savez, à produire un comté de qualité. La filière comté est l’une des plus vertueuses au monde : c’est du moins ce que dit

Par cet amendement, le Gouvernement propose une rédaction que j’estime équilibrée. Il prévoit une révision du dispositif qui repose sur les principes suivants

Les référentiels liés aux agréments des entreprises comporteraient des points de contrôle, qui garantiraient la qualité du conseil. De plus, l’exercice de l’activité de conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques resterait interdit aux fabricants de ces produits, compte tenu du risque élevé de conflits d’intérêts. Ainsi, les règles de séparation capitalistique des activités de conseil et de vente continueront de s’appliquer pour les producteurs de produits phytopharmaceutiques.

prévenir les conflits d’intérêts. Cela concernera un secteur bien particulier, une situation bien particulière

Mme la ministre.

l’activité de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques resterait interdite aux fabricants desdits produits. Cet élément a son importance. En tout état de cause, on ne peut pas rester en l’état,

la séparation du conseil et de la vente pour les fabricants de produits phytosanitaires. Oui ! En revanche, nous avons supprimé la séparation du conseil et de la vente pour les distributeurs,

rapide pour produire tous les effets escomptés.

Vous le savez, ces certificats encouragent la diffusion des pratiques économes en produits phytosanitaires. Ce dispositif a été lancé en 2016, initialement sous la forme d’une expérimentation centrée sur les distributeurs. lorsque la loi Égalim les a pérennisés, le périmètre a été élargi à d’autres acteurs, à savoir les déclarants à la redevance pour pollutions diffuses. Cependant, l’élargissement du dispositif crée des difficultés, car ces acteurs ne disposent pas des leviers auxquels ont recours les distributeurs pour promouvoir des solutions alternatives et, donc, pour générer des certificats. En outre, ces acteurs ne représentent qu’une très faible proportion – 1 % – des obligations générées par le dispositif, essentiellement, d’ailleurs, dans les zones frontalières. Dans ce cadre, il me paraît nécessaire, comme le Gouvernement s’y est engagé, de procéder à une simplification administrative en recentrant le dispositif sur les distributeurs de produits phytopharmaceutiques.

Face à une telle volonté de dérégulation de l’usage des pesticides, y compris pour des produits interdits comme les néonicotinoïdes, ces insecticides tueurs d’abeilles, le rapporteur a lui même reconnu que le dispositif initial était contraire au droit européen.

à cette inversion des valeurs qui privilégie le nivellement par le bas de nos normes sanitaires et environnementales, je crois nécessaire de rappeler que ces interdictions de mise sur le marché sont ordonnées non pas pour entraver les travaux agricoles, mais pour protéger la santé des sols et, bien évidemment, celle des travailleurs de la terre.

Dépourvues de toute rationalité, la totalité des mesures figurant dans cet article sont une négation de l’impact des pesticides sur l’environnement. La parole est à M. Vincent Louault,

sur l’article. Cet article modifie le code de la santé publique et a des implications importantes, non seulement sur la procédure applicable aux produits phytopharmaceutiques, mais aussi dans de nombreux autres domaines.

pour le contrôle sanitaire des eaux, aux procédés de traitement des eaux, aux produits phytopharmaceutiques, aux fertilisants, aux produits biocides et aux additifs destinés à l’alimentation animale. Ce principe d’information préalable des tutelles de tout projet de décision pris au nom de l’État que vous souhaitez inscrire dans la loi est très préoccupant.

involontairement, à ne pas faire le distinguo entre les différentes formes de néonicotinoïdes. Un peu de pédagogie et d’éclairage scientifique me semblent importants, afin d’être le plus juste et le plus objectif possible. Les néonicotinoïdes

2021 et 2022. De nouvelles études toxicologiques ont encore eu lieu en 2023 et 2024. Dans une publication de janvier 2022, le groupe scientifique de l’AESA sur les produits phytopharmaceutiques et leurs résidus a conclu qu’il n’existait aucune preuve d’un risque plus élevé associé à l’acétamipride par rapport à l’évaluation antérieure en ce qui concerne la biodiversité, la génotoxicité, la toxicité pour le développement et la neurotoxicité, y compris la neurotoxicité développementale et l’immunotoxicité. L’AESA est parvenue à la conclusion que, d’une manière générale, les informations fournies ne démontraient pas que l’acétamipride était susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement. Rappelons que l’acétamipride est aujourd’hui utilisé

qui disposent que l’évaluation en vue d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit doit être indépendante, objective et transparente au regard des connaissances scientifiques et techniques actuelles. S’en remettre au ministre chargé de l’agriculture créerait un doute sérieux quant au respect de ces critères. Le fait de confier cette possibilité au directeur général de l’Anses constitue également un problème en soi, puisque l’on peut craindre que cela ne nuise à l’indépendance de l’évaluation, en cas de pression extérieure pour qu’il la délègue. Rien ne justifie cette mise sous tutelle. L’Anses rappelle elle même que son indépendance et celle de ses agents sont un critère essentiel de la qualité, de la légitimité et de la crédibilité de l’expertise scientifique qu’elle met en œuvre.

dans ces territoires, dès lors que toutes les garanties de sécurité pour l’homme et l’environnement sont réunies. Cependant, nous refusons que cela se fasse au détour d’une proposition de loi dépourvue d’étude d’impact, alors même que les dernières études de l’Anses démontrent que le bilan des expérimentations dans ce domaine reste très mitigé.

le sujet, et, il faut le rappeler, du nombre de dérogations votées ces dernières années. Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article, dont les dispositions déséquilibreraient fortement notre système actuel.

Du reste, le voudrais je que je ne le pourrais pas, tout simplement parce que les prérogatives du directeur général de l’Anses sont encadrées par des dispositions européennes

Merci

d’interminables débats, comme celui que nous allons avoir sur l’acétamipride. De même, cela éviterait les distorsions de concurrence résultant de surtranspositions.

Cet amendement ne revient aucunement sur l’indépendance de l’Anses, qui est garantie non seulement par la loi, mais aussi par le droit conventionnel. C’est la raison pour laquelle je vous propose

Il s’agit d’une démarche double : préserver la biodiversité et la santé publique tout en soutenant nos agriculteurs dans leur indispensable transition écologique. Les produits phytosanitaires conventionnels, bien qu’indispensables pour répondre à certains enjeux agricoles, posent des problèmes majeurs en matière de pollution des sols, des eaux et des écosystèmes. Ils impactent directement la biodiversité, mettant en péril les pollinisateurs essentiels à nos cultures, et affectent potentiellement la santé humaine. Pour relever ce défi, il est impératif que l’État prenne ses responsabilités en investissant massivement dans la recherche et l’innovation. Cela passe bien évidemment par le développement de solutions alternatives : biocontrôle, agroécologie, nouvelles techniques de lutte intégrée, soutien financier et technique aux agriculteurs. La transition vers des pratiques plus durables doit être non pas une contrainte insurmontable, mais une opportunité d’avenir, une approche proactive et collaborative impliquant agriculteurs, scientifiques et entreprises innovantes pour coconstruire des solutions adaptées aux réalités du terrain. Ce texte s’inscrit donc dans une vision à long terme : protéger nos ressources naturelles et nos territoires tout en garantissant la pérennité et la compétitivité de notre agriculture. L’innovation et la durabilité sont non pas des choix opposés, mais bien les deux piliers d’un avenir agricole prospère. Les deux

En matière de biocontrôle, un soutien annuel de 20 millions d’euros en moyenne est apporté par l’État à des projets de recherche et d’innovation conduits par des entreprises et des laboratoires de recherche, notamment dans le cadre du plan France 2030.

Seraient incluses dans le périmètre de cette obligation toutes les missions relatives aux médicaments vétérinaires, aux pesticides, aux produits biocides, à l’agrément des laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux ou encore aux additifs utilisés en alimentation animale. Il s’agit d’une remise en cause claire et nette de l’Anses et de son indépendance.

les dossiers d’AMM de produits phytopharmaceutiques. Or la rémunération qu’elle perçoit est bien inférieure aux coûts qu’elle supporte pour instruire ces dossiers, de plus en plus nombreux. Vous pourriez donc

Je vous remercie

et ce en deux décennies seulement. Entre 2011 et 2021, notre solde commercial agricole a chuté de 12 milliards à 8 milliards d’euros et nous importons désormais 50 % de ce que nous consommons, soit deux fois plus qu’en l’an 2000.

a montré ses limites. Si cette agence fournit un éclairage scientifique essentiel, elle ne prend pas en compte les enjeux économiques, commerciaux et stratégiques liés à ces autorisations. Cela crée des distorsions de concurrence avec nos partenaires européens et fragilise encore davantage notre agriculture. Cet amendement vise à redonner au ministère de l’agriculture la compétence de délivrance de ces autorisations, en s’appuyant sur les avis scientifiques de l’Anses, tout en assurant un arbitrage équilibré entre les impératifs sanitaires, environnementaux et économiques. et économiques. Il s’agit d’un choix de souveraineté et de pragmatisme pour permettre à notre agriculture de répondre aux défis d’aujourd’hui sans être pénalisée par les interdictions arbitraires. Ce retour au bon sens est indispensable pour garantir la compétitivité de nos agriculteurs, préserver notre autonomie alimentaire et réaffirmer le rôle stratégique du ministère de l’agriculture.

sur les situations dans lesquelles des contraintes techniques rendent impossible le traitement par voie terrestre. Il s’agit notamment de prendre en compte la réalité du terrain dans les zones escarpées et difficiles d’accès, mais également la hauteur des parties végétales à traiter en arboriculture, qui fait obstacle à l’efficacité du traitement. Cet amendement vise à définir un cadre clair pour limiter au strict nécessaire la pulvérisation par drone, qui ne serait autorisée que lorsque les conditions techniques rendent impossible l’application terrestre sur les cimes des arbres les plus hauts, ou lorsqu’elle présente des avantages manifestes pour la santé et l’environnement.

de loi. Monsieur le président, madame la ministre,

Merci,

interdit l’utilisation des produits phytopharmaceutiques de la classe des néonicotinoïdes et assimilés en France. Cette interdiction avait été approuvée par le législateur en 2018. Il s’agissait à l’époque d’une surtransposition assumée par les parlementaires.

que « les limitations portées par le législateur à l’exercice de ce droit ne sauraient être que liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi

Merci,